a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Michel Durafour, qui fut sénateur de la Loire de 1965 à 1967 et de 1983 à 1988. Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 et de l'article 56 de la Constitution, la commission des lois a fait connaître qu'elle avait émis, lors de sa réunion du mercredi 2 août 2017, un vote favorable- 22 voix pour, 7 voix contre et 1 bulletin blanc -à la nomination de M. Michel Mercier aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel. félicitations à M. Mercier. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans la vie politique

Madame la présidente, il n'est nul besoin d'un long propos introductif pour saluer l'accord que nous avons obtenu en commission mixte paritaire sur les deux projets de loi,

à réduire à néant cette source de financement, comme si un combat était mené contre les communes rurales de ce pays, mais aussi contre un certain nombre d'associations,

Je voudrais vous dire néanmoins que l'accord trouvé sur le projet de loi ordinaire reprend un grand nombre des positions que vous avez adoptées, mes chers collègues,

Il est six points sur lesquels le Sénat a obtenu satisfaction dans la discussion en commission mixte paritaire. Il s'agit d'abord, pour plusieurs de ces points, de la symétrie que nous entendions imposer entre les obligations

les conditions, les modalités et les limites de leur prise en charge. Je suis très impatient de découvrir la teneur de ce décret. C'est ainsi que, sur l'initiative de notre collègue Collombat, nous avons maintenu

enfin, que s'agissant de la rémunération de collaborateurs à temps partiel par les, l'interdiction posée pour les parlementaires vaudra aussi pour les ministres, ce qui est bien le moins, compte tenu des responsabilités que ceux-ci exercent. Nous avons accepté, pour ce qui concerne l'inéligibilité liée à des crimes ou à des délits commis par un candidat à une élection, un amendement déposé à la toute dernière minute, puisque je l'ai découvert dans la nuit de lundi à mardi, faisant mention

que la peine d'inéligibilité prononcée par le juge, au moment où celui-ci condamne un prévenu à une peine liée à un crime ou à un délit, doit figurer dans le casier judiciaire. Cela va sans dire, vous le savez bien, puisque cette obligation existe déjà et qu'elle est du niveau réglementaire. Pour des raisons qui m'échappent, le Gouvernement a tenu à le préciser de la manière la plus nette qui soit dans la loi. C'est la position qu'a défendue mon homologue de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas voulu

de substance. Je le suppose, d'aucuns voudraient pouvoir dire que, ainsi, l'engagement du Président de la République d'empêcher l'accès à la fonction parlementaire de quelqu'un ayant une peine inscrite à son casier judiciaire aura été tenu. Tel n'est heureusement pas le cas, car, si cela l'avait été,

le condamné le demande, dans d'autres cas, il n'en ressent pas l'utilité, ce qui crée une inégalité entre Français condamnés à la même peine et pour le même délit ou le même crime. La peine d'inéligibilité, en revanche, prononcée par un juge du siège,

des investissements pour les petits équipements des communes que nous défendions et dont le Gouvernement n'a pas voulu. Nous ne manquerons pas de le rappeler à l'ensemble des maires de France

j'ai plaisir à me retrouver aujourd'hui devant vous, puisque vous êtes saisis des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la confiance dans la vie politique. Je tiens à saluer M. le président Bas, rapporteur de la CMP, qui a présenté les points d'accord ayant permis aux deux assemblées de converger sur le projet de loi ordinaire. Cela n'a pas été possible, monsieur le président, vous l'avez souligné, sur le projet de loi organique, que vous examinerez en nouvelle lecture après-demain.

le projet de loi ordinaire, chaque assemblée a pu faire un pas l'une vers l'autre, ce qui est pour moi un grand motif de satisfaction. C'est dans ce genre de circonstance que l'on mesure réellement ce qu'est un travail parlementaire constructif, effectif, fondé sur des convictions solides de part et d'autre, mais aussi sur le respect et l'écoute mutuels, donc sur la volonté de légiférer positivement. Tout d'abord, plusieurs dispositions qui, pour le Gouvernement et l'Assemblée nationale, paraissaient se situer hors du champ initial de la réforme n'ont pas été réintroduites en CMP. Elles concernaient pour l'essentiel la fonction publique. Le Gouvernement avait fait valoir, suivi en cela par l'Assemblée nationale, que le périmètre originel du projet de loi n'incluait aucune thématique relative à la fonction publique. Nous avions également ajouté qu'une loi très récente, celle du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires, venait seulement d'entrer en vigueur et qu'il nous semblait plus pertinent d'évaluer les conséquences des dispositifs que cette loi proposait avant de légiférer à nouveau. Le Gouvernement avait défendu cette position, et la CMP n'a pas rétabli ce type de disposition. La CMP, vous l'avez souligné, monsieur le président, a toutefois adopté un article 2 E demandant au Gouvernement un rapport sur le remboursement des frais de scolarité pour les anciens élèves de plusieurs grandes écoles lorsque ceux-ci n'effectuent pas la totalité des années de travail qu'ils doivent au service de l'État. L'intérêt d'une disposition prévoyant la remise d'un rapport se rapportant à un sujet qui est déjà réglé par voie de décret n'est pas apparu déterminant au Gouvernement. Toutefois, bien entendu, nous prenons acte du choix qui a été effectué par la CMP. Il en est de même de deux autres dispositions. La première, vous l'avez rappelé, monsieur Bas, concerne les frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement. Il semble au Gouvernement que cette disposition est surabondante, puisque, comme j'ai pu l'indiquer en première lecture, les dépenses liées aux fonctions ministérielles, telles que les frais de représentation ou de réception, sont déjà soumises au contrôle au contrôle que vous souhaitez voir instaurer, que ce soit par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère ou,, par la Cour des comptes. Quant à la création par décret en Conseil d'État d'un registre des déports pour les ministres, j'ai eu l'occasion de montrer que ces derniers étaient déjà soumis à un mécanisme rigoureux de déport par décret. Ce dispositif a d'ailleurs trouvé à s'appliquer pour l'actuel Gouvernement. La CMP a souhaité maintenir un tel mécanisme qui, de mon point de vue, pourrait poser des difficultés au regard du principe de secret des délibérations du conseil des ministres. Il appartiendra au Conseil constitutionnel, s'il est saisi, d'en apprécier la constitutionnalité, et et nous saurons qui, de l'un ou de l'autre, avait raison sur ce point. En toute hypothèse et au-delà de nos points de vue juridiques différenciés, le Gouvernement prend acte des dispositions qui ont été adoptées par la CMP et respecte évidemment sa volonté. L'essentiel,

Le premier point fort s'attache à l'inéligibilité des personnes qui commettent des crimes ou des délits. La commission mixte paritaire a repris le dispositif voté par les deux assemblées en le renforçant. La liste des délits conduisant à l'inéligibilité automatique, sauf décision contraire du juge, a été élargie, notamment en reprenant des propositions du Sénat. Comme la CMP l'a souhaité, faisant en quelque sorte la synthèse des débats parlementaires, ce qui est d'une certaine manière son office, il est désormais clairement prévu l'obligation pour tout prétendant à une élection de posséder un casier judiciaire B2 vierge de toute peine d'inéligibilité prononcée pour des crimes ou pour l'ensemble des délits qui sont visés par le texte que vous avez adopté.

Le deuxième point concerne la prévention des conflits d'intérêts pour les parlementaires. La définition du conflit d'intérêts est adaptée à la réalité du mandat parlementaire, et un mécanisme de déport est prévu dans le respect de l'autonomie des assemblées. L'interdiction des emplois familiaux apparaît également comme un point important du texte. Là encore, un accord s'est dessiné sans heurts entre les deux assemblées, au-delà d'une petite péripétie vite oubliée. C'est un acquis attendu par les Français, qui n'acceptent plus désormais une telle pratique. Parallèlement,

constituent, de ce point de vue, un socle solide pour progresser dans ce domaine. Le quatrième apport du texte tend à la suppression de l'IRFM et à la mise en place, M. le président Bas l'a rappelé, d'un mécanisme approprié de contrôle des frais de mandat des parlementaires. Nous avions déjà beaucoup progressé avec votre rapporteur lors de la première lecture, et c'était un motif de satisfaction, chacun, je crois, ayant compris les préoccupations de l'autre. La commission des lois de l'Assemblée nationale a approfondi le travail que nous avions engagé, aboutissant à à un accord qui me semble équilibré et qui, tout à la fois, introduit la rigueur des contrôles et garantit la souplesse de la mise en oeuvre nécessaire au fonctionnement de la vie parlementaire, dans le respect de l'autonomie des assemblées. Le projet de loi ordinaire prévoit aussi, et c'est le cinquième grand axe de ce texte, les conditions dans lesquelles le Président de la République et le Premier ministre peuvent, avant la nomination d'un membre du Gouvernement, vérifier qu'il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts, qu'il est en règle sur le plan fiscal et que son casier judiciaire B2 est vierge. Le texte B2 est vierge. Le texte ne concerne donc pas seulement les parlementaires, comme j'ai pu l'entendre trop souvent au cours des dernières semaines. Cette exigence avait été en particulier portée par votre rapporteur. Elle est désormais satisfaite. Le texte contient, enfin, des dispositions renforçant le contrôle des ressources des partis politiques et des candidats, ainsi que celui des prêts qui leur sont accordés. Parallèlement, avec le médiateur du crédit et la banque de la démocratie, sera facilité l'accès au financement bancaire des partis et des candidats, afin de renforcer le pluralisme de notre vie politique. Là encore, nous avons pu avoir des désaccords ponctuels, mais le texte adopté par la CMP est très satisfaisant. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, au-delà des débats, de la confrontation nécessaire et utile que nous pouvons avoir entre des points de vue politiques ou juridiques, nous avons pu observer un mouvement vers un objectif commun tendant à renforcer la confiance dans la vie politique. C'est le fruit d'une ambition partagée et des bonnes volontés que j'évoquais devant vous en première lecture. Votre rapporteur faisait d'ailleurs état, à ce moment-là, d'un mouvement fédérateur. Que le Sénat et l'Assemblée nationale aient pu s'accorder est, je crois, un signal positif pour nos concitoyens. Il témoigne de l'esprit de responsabilité des parlementaires, de leur volonté de répondre aux attentes des Françaises et des Français, qui appellent à plus de transparence et d'éthique dans les pratiques politiques. Au nom du Gouvernement, je tenais très sincèrement à vous en remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, en particulier M. Philippe Bas, votre rapporteur, qui n'a ménagé ni son temps ni son énergie pour aboutir à ce résultat positif, gage d'une confiance partagée.

Madame la présidente, monsieur le président et rapporteur, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la confiance entre les citoyens et leurs représentants, chacun ici en est conscient, est actuellement en crise. Les principaux symptômes de cette crise de confiance, qui ne touche pas uniquement notre pays, sont l'abstention, la désaffection pour les institutions et les élus, ainsi que la floraison de mouvements populistes et radicaux. Pour remédier à cette crise qui abîme notre démocratie, le Gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi « rétablissant la confiance dans l'action publique ». Les dispositions de ce texte avaient principalement pour objet de durcir le régime de l'inéligibilité en cas de manquement à la probité, de fixer un cadre aux conditions d'embauche et de travail des collaborateurs d'élus, en interdisant notamment les emplois familiaux, de réformer les conditions de rémunération des parlementaires et de renforcer la lutte contre les conflits d'intérêts et le contrôle du financement de la vie politique. Le projet de loi, désormais intitulé « pour la confiance dans la vie politique », après avoir été examiné par la commission mixte paritaire, est une nouvelle fois soumis à notre assemblée. Malgré son objet particulier, de loi a été discuté et adopté par le Parlement dans de bonnes conditions, ce dont chacun d'entre nous peut, à juste titre, se réjouir. Le texte final adopté mardi dernier par la commission mixte paritaire comporte un certain nombre des modifications que le Sénat avait apportées, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. nos amendements visant à donner aux assemblées une plus grande souplesse dans la gestion et la prise en charge des frais de mandat ont été, en substance, maintenus. Le système actuel de l'IRFM ne pouvait rester en l'état, mais il fallait absolument veiller à ne pas mettre en place une usine à gaz administrative, qui aurait produit des dépenses publiques nouvelles et des complexités inutiles. Sur les dispositions relatives à la peine complémentaire d'inéligibilité en cas de crimes ou de manquements à la probité, les apports du Sénat ont aussi été préservés. Cela ne peut faire oublier qu'un certain nombre d'amendements de bon sens votés par le Sénat ne figurent pas dans le texte final. Je pense notamment à l'ouverture des concours internes aux collaborateurs parlementaires, ou encore à la levée du « verrou de Bercy à souligner le fait que les dispositions relatives aux conditions d'emploi des collaborateurs d'élus, si elles constituent un progrès incontestable, ne sont pas suffisantes en l'état : un véritable statut des collaborateurs reste donc à créer. Au-delà de ces points particuliers, on ne peut que déplorer le caractère profondément lacunaire du texte, qui selon nous réduit son ambition première et nuit gravement à son efficacité. En effet, il est regrettable que le Gouvernement se soit borné à traiter du seul cas des parlementaires et des élus locaux. La crise de confiance que j'ai évoquée touche non pas uniquement le Parlement et les collectivités, mais aussi la haute fonction publique, la presse et le monde syndical. Pour qu'une action de rétablissement de la confiance puisse réussir, il aurait été indispensable de prévoir également des mesures fortes de transparence dans ces sphères de la vie publique. Tel n'a pas été le cas, et le Gouvernement a préféré se focaliser sur quelques sujets particuliers. La volonté du Gouvernement, comme du Parlement, de rétablir la confiance avec les citoyens n'est pas à remettre en cause ; elle s'est d'ailleurs traduite par un fort investissement de l'ensemble des acteurs et par une discussion parlementaire qui fut riche, mais hélas trop restreinte. Enfin, je tiens à dire un mot sur le projet de loi organique examiné conjointement par la commission mixte paritaire. Celle-ci, vous le savez, mes chers collègues, n'est pas parvenue à un accord sur le texte, les discussions ayant achoppé notamment sur la question de la réserve parlementaire. Nous regrettons profondément l'attitude des représentants de la majorité à l'Assemblée nationale concernant la question de la réserve parlementaire, et jugeons que leur attitude rigide et leur surdité aux arguments et aux propositions alternatives du Sénat sont tout à fait contraires à l'esprit d'écoute réciproque et de conciliation qui doit présider au cours des commissions mixtes paritaires. Madame la garde des sceaux, c'est avec plaisir que mon groupe votera en majorité en faveur du projet de loi, mais cela ne doit pas faire oublier que celui-ci est en l'état insuffisant

qui doivent pouvoir bénéficier d'un délai et de conditions favorables pour trouver une autre activité.

Pour ce qui est des apports plus spécifiques du Sénat, mes chers collègues, je veux évoquer la question des collaborateurs parlementaires. En effet, il eût été choquant

En ce qui concerne la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité, madame la garde des sceaux, on nous a beaucoup rappelé, hier matin,

Nous en avons beaucoup parlé, mais il existe toujours, à la fin de ce débat, 451 partis politiques en France. La question, certes complexe,

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, je voudrais tout d'abord rendre hommage à M. Bas, notre président et rapporteur, que je considère comme un grand connaisseur de la Loi, avec une

accord ait été trouvé en CMP sur ce projet de loi ordinaire. Si ce texte comprend de nombreuses avancées, nous restons quelque peu dubitatifs sur son impact final, une fois qu'il sera entré en application. ce n'est pas seulement par une prétendue moralisation que l'on rétablira la confiance. Nos concitoyens attendent aussi davantage d'éthique. Et nous devons continuer à faire nôtres certaines règles de déontologie. Veillons à ce que l'antiparlementarisme ambiant et la précipitation ne nous empêchent pas de légiférer sur les véritables dangers susceptibles de menacer le principe fondamental de la séparation des pouvoirs.

Avec ce dispositif controversé, on s'expose à de nouvelles affaires politico-financières qui renforceront la défiance de nos concitoyens à l'égard des politiques, malgré le vote de cette loi de prétendue « moralisation »- un un mot qui me fait peur ! En revanche, nous sommes satisfaits de l'élargissement du champ des infractions pouvant conduire à une peine d'inéligibilité : délits de harcèlement et de violences sexuelles, provocation à la haine en raison de la race, du sexe ou de l'orientation sexuelle. Cela étant, et n'en déplaise aux sénateurs du groupe La République en marche, la confiance s'obtient d'abord en sachant tenir ses engagements de campagne. Il reste encore beaucoup à faire pour rétablir le lien de confiance avec nos concitoyennes et concitoyens, en dépassant nos intérêts politiques immédiats, en renonçant aux postures et en nous montrant davantage en empathie avec elles et avec eux, bien sûr sans tomber dans le populisme anti-politiciens, anti-médias, anti-fonctionnaires et presque « anti-tout actuellement en vogue, alimenté par l'extrême droite, que nous avons déjà connu dans le passé avec le poujadisme et qui dessert le fonctionnement de la démocratie, en caressant les mauvais penchants des uns et des autres. Bravo

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, à l'issue d'une commission mixte paritaire qui a conclu, nous sommes saisis d'un texte amélioré et complété, répondant aux objectifs assignés par le Gouvernement. C'est le résultat d'un bon dialogue, à l'intérieur de chaque assemblée et entre les deux assemblées-

Il n'est donc pas surprenant que le sens de nos travaux soit peu lisible pour les citoyens et que les complaintes se multiplient sur la prolifération législative. Nous devrons,

qui nous conduisent, y compris lorsque l'un des nôtres a franchi de façon patente les limites de la décence élémentaire, à faire comme si rien ne s'était passé.

Ce sera, me semble-t-il, la meilleure réplique aux surenchères de ceux qui font profession de démolir tout titulaire d'un pouvoir issu de la démocratie.

aujourd'hui, nous concluons l'examen du projet de loi ordinaire et, vendredi prochain, nous reviendrons pour le projet de loi organique. Ce sera une curieuse façon de célébrer le 228 anniversaire de la nuit du 4 août 1789, qui a aboli les privilèges et fait disparaître les archaïsmes, surtout quand on sait comment s'est conclue la CMP sur le projet de loi organique, notamment au sujet de la réserve parlementaire parlementaire ! Pour nous, le problème, ce n'est pas que les parlementaires travaillent et que la session s'allonge, c'est que le Gouvernement choisisse le coeur de l'été pour s'exonérer du contrôle de l'opinion publique sur un sujet qui nous paraît très important. Après un examen précipité et souvent chaotique, nous sommes donc aujourd'hui parvenus à la fin du processus législatif sur ce projet de loi ordinaire qui traite de probité et d'exemplarité des élus. cette exigence est juste et nécessaire, impérieuse même, ce texte, malheureusement, n'est qu'un énième coup d'épée dans l'eau : la portée de ses mesures n'est pas à la hauteur des enjeux, et le système libéral continue de répandre de l'immoralité dans notre société. L'indécente plus-value de la ministre du travail à l'orée d'un plan social chez Danone jette gravement l'opprobre sur nos travaux et sur la légitimité de ce gouvernement à ériger la confiance comme modèle d'action politique. Je ne reviendrai pas ici sur les multiples démissions gouvernementales, toutes dues à ce qu'on appelle pudiquement « les affaires », mais je reste malheureusement persuadée qu'il faudra plus que ce texte pour ramener le peuple vers la le peuple vers la politique. Le désamour entre un peuple et ses représentants ne vient pas principalement de ce que sont ces derniers, mais du système lui-même, qui permet que le pouvoir soit capté par une élite, qui permet que la politique soit asservie aux intérêts de la finance mondialisée. Un pouvoir qui n'est pas guidé par l'intérêt général et la réponse aux besoins, mais par d'autres objectifs relevant d'intérêts privés. Le nouveau Président de la République, fraîchement sorti de l'ENA, repéré lors des travaux de la commission Attali pour devenir banquier d'affaires avant de revenir dans les allées du pouvoir, symbolise à lui seul le mélange entre intérêt privé et public. Argent et pouvoir font toujours bon ménage. Alors oui, les gens n'y croient plus, et que leur dire ? Depuis des décennies, la confiance est ébranlée par la parole non tenue, par les promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Les rendez-vous électoraux sont des mascarades de démocratie où la puissance de l'argent défend ses intérêts, que ce soit par la voie des médias dont elle est propriétaire ou encore par le financement des campagnes électorales. toujours les mêmes politiques qui sont menées, à rebours des intérêts populaires, alimentant le bataillon des abstentionnistes. Une politique de classe, où la démocratie est réduite à portion congrue, où les efforts sont demandés aux plus fragiles, comme c'est le cas avec la baisse des APL, les aides personnalisées au logement,

Tant que la politique ne permettra pas de dessiner un « en commun » pour l'ensemble de nos concitoyens, un projet fondé sur la possibilité d'un progrès partagé, on continuera d'alimenter la défiance et la colère. C'est malheureusement inévitable. Nous regrettons donc le contenu limité de ce texte, qui se résume en quelques mesures dont le relent antiparlementariste est assez déplaisant. Ce serait tellement plus facile de réduire le Parlement à un rôle de godillot de la majorité présidentielle, ou de faire en sorte qu'il écrive la loi et contrôle le Gouvernement dans les sous-sols ou dans les greniers,

Notre premier regret est donc celui d'une loi qui n'a pas de souffle, d'une loi de réaction aux affaires. Les emplois familiaux pour Fillon, le mensonge pour Cahuzac, la phobie administrative pour Thévenoud Oui, de telles situations ne doivent plus se reproduire. Ces quelques mesures sont donc évidemment positives, mais aussi profondément lacunaires. Pourquoi ne pas avoir accepté de faire sauter le « verrou de Bercy », comme nous l'avions fait adopter en première lecture au travers d'un amendement ? Voilà un élément de confiance qui permettrait de lutter contre la délinquance financière au plus haut niveau. Avec cette loi, les évadés fiscaux continueront de dormir tranquilles. Deuxième regret, le détricotage des avancées du Sénat pour limiter les pratiques du pantouflage et pour cesser les conflits d'intérêts au sein de la haute fonction publique. Il reste un vague rapport rapport ... Ce recul est un aveu ! Heureusement, la CMP a réintégré les propositions du Sénat pour soumettre aux mêmes règles de déontologie les membres du Gouvernement. C'est un minimum. Troisième regret, toute velléité de moraliser les médias ou la vie économique a été balayée d'un revers de main, alors que, pour nous, confiance, démocratie et justice sociale vont de pair. Les enjeux de démocratisation de nos institutions ont été balayés d'un revers de main : la proportionnelle, le droit de vote pour les étrangers, un droit de pétition renforcé, la création d'un statut de l'élu. Nous pensons que le problème de confiance vient aussi du manque de représentativité de nos institutions. Nous sommes satisfaits du début de reconnaissance d'un statut pour les collaborateurs parlementaires, parlementaires, même si nous aurions pu aller plus loin en reconnaissant des passerelles, comme nous l'avions fait adopter en première lecture. Nous serons très attentifs aux déclinaisons réelles de ces articles. Pour autant, nous sommes inquiets de la disposition qui vise à faire connaître aux organes de déontologie les fonctions politiques de nos collaborateurs. À partir du moment où il s'agit de fonctions non rémunérées, une telle disposition constitue, selon nous, une atteinte aux libertés individuelles et au respect de la vie privée.

en croire François Bayrou, son initiateur, l'objet de la grande loi de moralisation dont il s'était fait le propagandiste était d'empêcher que les intérêts privés, financiers et industriels prennent en otage » la vie publique de notre pays. Au terme de débats montrant qu'il ne suffisait pas de changer le personnel politique pour améliorer le parlementarisme, que reste-t-il de cette belle ambition ?

de déclarations, autant de tracasseries et d'occasions de contentieux pour les élus et les responsables politiques. Un « libéralisme bureaucratique », tel est la spécificité française, avec quelques autres particularités comme le « favoritisme institutionnel inversé » : si j'embauche mon épouse comme assistante, je commets un délit,

On ne peut pas parler d'un progrès considérable ! Je pourrai continuer longtemps, tant les obligations contraignantes, mais sans réelle portée, sont nombreuses dans les deux textes. Quant aux dispositions relatives au financement de la vie publique, il était difficile de faire plus compliqué pour un résultat aussi modeste. revanche, s'agissant de l'essentiel, c'est-à-dire de la prise en otage de la vie publique par les grands intérêts privés ou de la porosité de plus en plus grande entre la nébuleuse politique qui gravite autour du consul présidentiel, la haute bureaucratie d'État et les milieux d'affaires,

a expliqué qu'essayer de limiter le pantouflage reviendrait à empêcher « la fluidification d'affectations successives entre secteur public et secteur privé rendrait difficile le recrutement de personnes ayant développé des compétences dans le secteur privé sur des emplois [ ...] en lien avec ces compétences.

de sortir le pays de la stagnation que la thrombose financière a laissée, de contenir l'évasion fiscale ou de redonner à la France l'assise industrielle qu'elle a perdue ? J'ai cherché et je n'ai pas trouvé Moralisez, moralisez, il en restera toujours quelque chose, mais certainement pas une plus grande confiance dans la vie publique ou politique. Tout au contraire, se plier au vent démagogique ne fera que donner du grain à moudre à la campagne anti-élus qui, depuis des années, sert de cache-misère aux échecs des exécutifs qui se sont succédé. La société de cour qu'est devenue l'arène politique française a remplacé le débat par la lapidation médiatique. Déclenchée Déclenchée au bon moment, celle-ci permet de se débarrasser d'un concurrent gênant ou de forcer la décision. Consolation : le retour de flamme est rarement loin

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, chers collègues, lors de son audition au Sénat, Mme la ministre a évoqué la nécessité d'un « choc de confiance » dans notre vie politique : un choc de confiance qui prendrait la forme, selon les auteurs de ce projet de loi, de l'introduction d'une multitude de nouvelles dispositions en matière de probité et d'éthique pour les élus. Une telle proclamation a de quoi surprendre, si l'on se souvient de la trentaine de textes qui ont été votés précédemment et qui ont imposé de nouvelles exigences aux responsables publics. Nous-mêmes avons pris nos responsabilités dans cette assemblée, avec notre comité de déontologie parlementaire, instrument du respect d'une certaine règle de conduite.

Le Sénat a accueilli le projet de loi initial avec une grande vigilance. Il a toujours porté une attention particulière au respect de la Constitution, des libertés et des droits fondamentaux, en particulier la liberté de candidature, la liberté de fonctionnement des partis politiques et la séparation des pouvoirs. De même, le Sénat devait s'assurer que les collectivités de toutes tailles ne soient pas astreintes à d'injustes sacrifices. Je pense en particulier à la réserve parlementaire, dont la suppression, que j'évoquerai ultérieurement, aura des conséquences néfastes sur les projets de nos communes. Ce texte a manifestement été rédigé dans la précipitation. Le Sénat a néanmoins fait preuve d'ouverture d'esprit et a souhaité apporter sa contribution de législateur et de défenseur des élus locaux. grâce à l'esprit de discernement de notre président et rapporteur, le Sénat a comblé un certain nombre de lacunes. Je pense notamment au renforcement des garanties pour les collaborateurs familiaux qui seront licenciés par l'effet « couperet » du présent texte. Nous leur devions d'améliorer leur sort, car ils travaillent dans le sens de l'intérêt général. Ils vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans leur transition professionnelle, ainsi que de délais plus adaptés que ceux qui avaient été initialement prévus. Nous avons introduit dans le texte un dispositif sûr et réaliste pour la gestion des frais de mandats et des indemnités parlementaires, dans le respect de l'autonomie des assemblées, afin de permettre un contrôle efficace. J'ajoute que nous avons veillé à élaborer un texte qui rétablisse la confiance à l'égard de l'ensemble des acteurs de la vie publique : élus, certes, mais aussi membres du Gouvernement et fonctionnaires. Mes chers collègues, les exigences en matière de bonne conduite et de transparence s'appliquent à tous. Le texte du Gouvernement était, à cet égard, particulièrement lacunaire et d'une discrétion de violette, sans doute due à une trop grande modestie ou à un altruisme trop exclusif. Aussi, sur l'initiative de notre groupe, le Sénat a introduit un nouveau titre relatif à la déontologie des fonctionnaires. Le législateur doit s'emparer de la question des allers et retours de certains hauts fonctionnaires ou agents publics en disponibilité, entre la fonction publique et le secteur privé, qui laissent perplexes beaucoup de nos concitoyens. C'est ainsi que le texte adopté par le Sénat prévoyait plusieurs dispositions, dont des délais de carence pour encadrer les retours du secteur privé vers la fonction publique. Malheureusement, ce titre entier, et on comprend mal pourquoi, n'a pas survécu à l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Le Sénat a créé un registre des déports pour les ministres confrontés à un conflit d'intérêts en conseil des ministres et prévu qu'un décret définirait les conditions de prise en charge des frais de représentation des membres du Gouvernement. Nous nous réjouissons que ces dispositions aient finalement été reprises par l'Assemblée nationale et acceptées par le Gouvernement. Nous avons aussi oeuvré pour préserver les droits de nos concitoyens concernés par cette loi, puisque le texte adopté par le Sénat fait défense aux membres du Gouvernement d'adresser à l'administration des impôts des instructions dans des affaires individuelles, dans le cadre de la délivrance de l'attestation fiscale. Nous avons également supprimé un dispositif bancal et redondant, la « Banque de la démocratie », dont l'office envisagé est déjà largement rempli par les établissements de crédit. Enfin, le Sénat s'est montré particulièrement attentif au sort des collectivités locales qui, avec la suppression de la réserve parlementaire, verront immanquablement leurs ressources et leurs moyens d'action encore amputés, alors même qu'elles sortent affaiblies d'un régime drastique, puisque, sous le précédent quinquennat, un effort de 11 milliards d'euros leur a été demandé. Pour les cinq ans à venir,

rigoureux ! Nous avions proposé, à titre de substitution, un fonds dédié et la participation de tous les parlementaires, de droit, aux commissions attribuant la DETR, la majorité gouvernementale, engoncée dans ses promesses de circonstance, n'a pas retenu nos propositions. De manière générale, le Gouvernement a été très sélectif dans la reprise des apports du Sénat, préférant une vision parfois étriquée- j'allais dire « climatique » -qui est de nature, en fin de compte, à affaiblir les élus. Ainsi, à l'issue d'un examen au déroulement tumultueux, l'Assemblée nationale est largement revenue sur plusieurs mesures clefs adoptées par notre assemblée. Bien plus, l'Assemblée nationale a supprimé l'intégralité du titre relatif à la à la déontologie des fonctionnaires. On comprend que l'intention du Gouvernement et de sa majorité est de poursuivre une démarche de mise à l'index, en refusant des règles de conduite qui s'imposeraient à l'ensemble des acteurs de la vie publique. Je note toutefois que la commission mixte paritaire réunie hier a fait preuve de plus de sagacité, choisissant de retenir plusieurs apports utiles du Sénat dont, notamment, la création d'un registre des déports pour les membres du Gouvernement et l'encadrement des frais des ministères.

Madame la présidente, madame la ministre de la justice, garde des sceaux, monsieur le président et rapporteur de la commission des lois, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier sincèrement les collègues

transparent, encadré par le ministère de l'intérieur, qui sert exclusivement à soutenir des projets d'investissements portés essentiellement par des communes rurales. Comme je l'avais indiqué le 10 juillet dernier dans le cadre de la discussion générale, depuis de nombreuses années, différents textes ont été adoptés, concernant par exemple la mise en place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les déclarations de patrimoine, la lutte contre les conflits d'intérêts, etc. Le dévouement des élus locaux

le contrôle des frais liés à l'exercice du mandat parlementaire et l'interdiction des emplois familiaux, la prévention des conflits d'intérêts,

Madame la présidente, madame la garde Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, depuis trente ans, trente lois ont été adoptées visant à prévenir, à supprimer et à sanctionner les pratiques qui entachent la vie politique. Une loi par an

Pourtant, si l'on considère les derniers mouvements de l'opinion, ces avancées n'ont pas suffi pour combler l'abîme de défiance qui sépare les citoyens des responsables publics, et plus particulièrement des parlementaires.

n'exclut pas tout contrôle », comme le disait Lénine, la politique impose des résultats. Ce à quoi Jaurès répond : « La République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. C'est bien là qu'est notre défi ! Oui, ce rejet de l'élu, c'est aussi le cri de colère d'un peuple orphelin, le résultat de promesses non tenues et d'espoirs déçus d'année en année. Avant tout texte de loi, il est du devoir de tout élu de la République d'être digne du pacte de confiance qui le lie à ses électeurs, cet acte dont parle Jaurès et dont la vitalité aujourd'hui est complexe. Cette confiance, elle vit chaque jour, dans cette assemblée, dans nos mairies ; la maintenir, voilà notre responsabilité d'élus

difficile de critiquer l'encadrement des activités de conseil et la vérification de la situation de la déclaration de patrimoine en fin de mandat pour le Président de la République. Sur le casier judiciaire, en revanche, les députés n'ont pas pris le risque d'adopter une disposition qui aurait pu être prétendument frappée « d'inconstitutionnalité Dommage que cette mesure phare du projet présidentiel, puis législatif, n'ait pas fait l'objet d'une analyse juridique en amont ! Du temps aurait été gagné et des illusions épargnées. chose est certaine : grâce à ces deux lectures, les Français auront pu juger de l'intérêt du bicamérisme. Oui, celles et ceux qui ont regardé la semaine dernière les débats en séance publique à l'Assemblée nationale et leurs couacs en série ont pu mesurer la nécessité du Sénat et de son travail. Un texte considéré unanimement par les observateurs comme enrichi et amélioré a été voté au Sénat, renforçant la lutte contre les conflits d'intérêts et pour la transparence, encadrant les emplois de collaborateurs parlementaires ainsi que les conséquences de leur licenciement en fin de mandat par leur « parlementaire-employeur ». Que les représentants associatifs et syndicaux des collaborateurs soient d'ailleurs également félicités pour leurs actions en la matière. Nous avons tous aussi pu déplorer, ici, le refus de supprimer le fameux « verrou de Bercy ». Outre ce point, le texte sénatorial limitait les conflits d'intérêts pour les hauts fonctionnaires et encadrait strictement cette pratique que l'on nomme « pantouflage » : bref, nous allions bien au-delà des intentions gouvernementales. Avec la version « allégée » du texte arrivée en séance au Palais-Bourbon, l'impression globale est double : de la précipitation et un ensemble sans grande cohérence. Un texte renommé au passage confiance dans la vie politique », histoire de souligner que l'homme malade de notre démocratie est bien l'élu, de préférence nanti de plusieurs mandats, et non le hiérarque de Bercy ou l'énarque oscillant entre secteur privé et secteur public. Pendant ce temps, les fonctionnaires « d'en bas » subissent dans nos hôpitaux, nos écoles et ailleurs des restrictions budgétaires et des conditions de travail déplorables, alors qu'ils concourent chaque jour au service public ! On a préféré s'attaquer à l'écume plutôt qu'à la vague, à certains petits arrangements plutôt qu'aux corrupteurs, livrer à la le cadavre de la réserve parlementaire plutôt que légiférer sur le casier judiciaire vierge des élus. Finalement, il y a surtout un vrai problème d'articulation juridique : c'est cette fameuse réforme institutionnelle que l'on nous annonce pour la rentrée

afin de permettre à la juridiction de déroger au prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité dans tous les cas prévus par cet article, tant pour les crimes que pour les délits, conformément à l'intention

Les amendements présentés par le Gouvernement en fournissent l'illustration : certains ont été approuvés par la commission, d'autres ont été sollicités

ce n'est pas une réponse claire et équitable pour les Français qui, eux, sont contraints de présenter un casier vierge pour toute candidature à plus de 350 professions. Comment le leur expliquer ?

du « verrou de Bercy » ? L'Assemblée nationale a rétabli ce que le Sénat avait supprimé à l'unanimité. Comment expliquer aux Français ce scandale du monopole du ministère de l'économie et des finances, cette exception au droit pénal français ? Une fois de plus, le Gouvernement et la majorité parlementaire qui a voté contre ces mesures fortes se sont placés au-dessus du peuple, au-dessus de la transparence et de l'éthique qui nous sont demandées. À chaque élu de s'appliquer désormais des règles d'exemplarité que ce texte n'aura pas su imposer.

chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, un mois après la présentation en conseil des ministres du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, la commission mixte paritaire chargée de l'examen de ses dispositions restant en discussion s'est réunie lundi à l'Assemblée nationale. Première CMP de la législature, elle a abouti à un accord. Je tiens, à cette occasion, à saluer la qualité du travail réalisé avec les députés, et notamment avec le rapporteur de la commission des affaires sociales, Laurent Pietraszewski. Loin de toute considération doctrinaire, nous sommes parvenus à rapprocher les positions de nos deux assemblées. Conscients de la nécessité de faire aboutir ce texte dans les meilleurs délais pour permettre au Gouvernement de se consacrer pleinement à la rédaction des ordonnances, nous avons adopté un texte de compromis, qui conserve néanmoins l'essentiel des apports du Sénat. Toutefois, et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à mes collaborateurs, n'oublions jamais ce que disait René Char L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant ». Très bien ! Vous le savez, nous approuvons la philosophie de ce texte, qui s'inscrit dans la continuité des travaux menés par notre assemblée depuis 2014. Ce projet de loi ne répond pas néanmoins à toutes nos attentes. En effet, il laisse de côté plusieurs sujets essentiels tels que la fixation par accord de la durée hebdomadaire de travail ou l'assouplissement du temps partiel et des seuils sociaux. Nous n'avons pas pour autant souhaité les introduire dans ce texte afin de rester dans le périmètre des habilitations demandées par le Gouvernement. Les travaux du Sénat ont donc visé à encadrer et à préciser ces dernières à travers l'adoption en commission, puis en séance publique, de 68 amendements. Ainsi, à l'article 1, nous avons prévu un motif spécifique pour tout licenciement d'un salarié qui refuse l'application d'un accord collectif. En CMP, nous avons précisé que ces salariés bénéficieront de droits renforcés à la formation. Soucieux de développer le dialogue social dans les petites entreprises dépourvues de délégué syndical, nous avons par ailleurs invité le Gouvernement à définir de nouvelles modalités pragmatiques de conclusion des accords collectifs, sans méconnaître les prérogatives des organisations syndicales. En outre, le texte adopté en CMP mentionne explicitement la possibilité pour l'employeur, comme le Sénat l'avait proposé, d'organiser une consultation des salariés pour valider un accord, tout en reconnaissant ce même droit aux organisations représentatives dans l'entreprise. Si nous nous sommes montrés très favorables à la création d'une instance unique de représentation du personnel à l'article 2, nous avons souhaité préciser ses règles de fonctionnement. Nous avons ainsi fixé à trois le nombre maximal de mandats successifs des représentants du personnel, sauf exceptions prévues par la loi, tout en renforçant leurs droits à la formation. Nous avons également veillé à garantir la transparence de ses comptes et soumis le recours à l'expertise à une mise en concurrence préalable. En CMP, nous avons confirmé la possibilité de créer en son sein une commission spéciale chargée des questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail afin de garantir la protection de la santé des salariés. À l'article 3, le point le plus débattu a été celui du périmètre géographique du licenciement économique. Le texte adopté par la CMP, fidèle à nos travaux, pose comme principe que la cause économique d'un licenciement devra désormais s'apprécier dans un périmètre national lorsqu'une entreprise appartient à un groupe international. Autrement dit, l'employeur, sous le contrôle du juge, devra justifier du motif économique du licenciement envisagé à l'aune de la situation des entreprises du groupe situées en France et relevant du même secteur d'activité. Nous avons toutefois laissé au Gouvernement la possibilité de déterminer d'éventuels aménagements à ce principe, ... Très bien ! ... et de retenir, par exemple, le périmètre de l'entreprise en cas de cessation d'activité, voire de redressement ... Très bien ! ... ou de liquidation judiciaire. Notre assemblée avait également invité le Gouvernement à mieux prendre en compte les besoins des travailleurs handicapés. Ainsi, nous avions prévu que les personnes handicapées devront avoir accès au futur site d'information sur le droit du travail. L'instance unique devra, en outre, être mieux associée aux décisions de l'employeur en matière d'emploi des personnes handicapées. Nous avions, par ailleurs, souhaité qu'ils bénéficient du développement du télétravail. Ces apports n'ont, fort heureusement, pas été remis en cause en CMP, tout comme les dispositions introduites au Sénat sur l'initiative du Gouvernement. Je pense notamment à la sécurisation des transferts conventionnels, à l'abaissement de l'ancienneté minimale d'un an pour bénéficier des indemnités légales de licenciement, ou encore à l'adaptation des règles relatives aux travailleurs détachés. Enfin, à l'article 9 portant sur le report de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, la CMP a conservé l'apport du Sénat exigeant que des analyses complémentaires sur les options alternatives soient remises par le Gouvernement avant la présentation du projet de loi de finances pour 2018, afin que que le Parlement dispose de tous les éléments d'information utiles pour statuer sur le devenir de cette réforme. J'en viens maintenant aux amendements adoptés par le Sénat qui n'ont pas été conservés en CMP. Tout d'abord, le Gouvernement pourra finalement harmoniser le régime juridique des accords de maintien de l'emploi, les fameux AME, avec celui des autres accords de flexisécurité. Vous le savez, madame la ministre, nous demandons la suppression des AME, dont l'échec est consommé, et qui ont perdu leur raison d'être depuis la création des accords de préservation et de développement de l'emploi par la loi Travail. Nul doute que la prochaine étape, une fois l'ordonnance publiée, sera leur abrogation. La CMP a ensuite rétabli l'habilitation autorisant le Gouvernement à aménager le calendrier de la généralisation des accords majoritaires. J'attire votre attention, madame la ministre, sur les dangers qu'une accélération de ce calendrier pourrait entraîner, en bloquant le dialogue social dans les entreprises. Si le Sénat est favorable aux accords majoritaires, il convient de faire précéder toute modification du calendrier de leur déploiement par des évaluations. Personne ne connaît en effet aujourd'hui la représentativité moyenne des syndicats signataires des accords collectifs, pas même, et je le regrette, vos services, madame la ministre. Il serait donc pour le moins paradoxal que ce texte, qui promeut avec raison la négociation d'entreprise, conduise à une diminution du nombre d'accords signés. La CMP est également revenue sur l'attribution de plein droit, sauf accord majoritaire contraire, de la compétence de négociation à l'instance unique. En effet, le texte prévoit désormais que cette instance pourra négocier des accords seulement si les partenaires sociaux dans l'entreprise l'y autorisent. Je reste toutefois persuadé que la compétence de négociation s'imposera d'elle-même dans quelques années, lorsque l'instance unique aura été mise en place dans toutes les entreprises. Le rétablissement de l'habilitation relative à la représentation des salariés dans les organes de gouvernance des grandes entreprises a également été voté. Le texte prévoit toutefois deux garde-fous pour tenir compte des observations du Sénat : d'une part, les seuils actuels d'effectifs ne seront pas modifiés ; d'autre part, l'ordonnance devra se limiter à améliorer la formation des représentants des salariés. En tout état de cause, une évaluation préalable des dispositions adoptées depuis 2013 est nécessaire avant de bouleverser de nouveau ce mécanisme. Nous avons bien compris le souhait du Gouvernement de se voir accorder certaines habilitations pour faciliter la négociation avec les partenaires sociaux, d'utiliser l'intégralité de ces habilitations, ou de n'y recourir qu'avec parcimonie, afin de ne pas alimenter l'instabilité juridique, dont nous souffrons tant déjà. Enfin, la CMP n'a pas souhaité fixer d'objectif précis à la réduction des délais de recours en cas de rupture du contrat de travail, tout en souhaitant à terme leur harmonisation. Madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous nous apprêtons à adopter porte la marque du Sénat, qui a été fidèle à ses convictions, tout en cherchant à accompagner le Gouvernement, dans un esprit de responsabilité. La majorité des sénateurs souhaite le succès de cette réforme, indispensable pour adapter notre droit social aux évolutions de notre économie et aux attentes des employeurs et des salariés. Nous n'avons pas le sentiment d'avoir préempté les résultats de la négociation avec les partenaires sociaux, qui va se poursuivre jusqu'à la publication des ordonnances. Le Parlement doit en effet pleinement jouer son rôle de législateur s'agissant de la première réforme sociale du quinquennat. La démocratie politique ne saurait s'effacer devant la démocratie sociale, et je crois que le texte adopté en CMP démontre que nous pouvons conjuguer ces deux légitimités dans une société moderne et apaisée. de dire à nos collègues députés la complexité de l'art d'agir, de légiférer, y compris d'ailleurs pour une chambre d'apaisement, en citant une fois de plus René Char : « La beauté naît du dialogue, de la rupture du silence et du regain du silence

C'est ce qui a orienté notre réflexion et nos débats sur le projet de loi d'habilitation que je soumets à votre vote aujourd'hui. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce sont, et je m'en félicite, nos expériences individuelles et collectives qui fondent les décisions prises sur ce texte. Vous avez enrichi nos discussions de votre expérience accomplie d'élu, car vous êtes en permanence au contact de nos concitoyens, mais aussi de leurs représentants locaux, à l'écoute de leurs inquiétudes et de leurs attentes face à un monde en profonde mutation. Votre expérience de parlementaire, en particulier sous la précédente législature, où vous avez examiné plusieurs réformes du code du travail, a, en outre, permis d'apporter des éclairages techniques indispensables à la qualité de nos échanges. Je tiens à vous en remercier tout particulièrement.

dans des entreprises de tailles différentes et dans des secteurs d'activité divers, en France ou à l'étranger. C'est tout l'apport de l'alliage de la démocratie politique et de la démocratie sociale. Enfin, nos discussions étaient chargées, au bon sens du terme, de notre expérience collective dans le temps. C'est-à-dire de notre histoire et des valeurs de la République qui fondent notre modèle social. C'est dire aussi la conviction d'une majorité d'entre nous, vous l'avez rappelé, monsieur le président-rapporteur, de la nécessité nécessité de rénover profondément notre modèle social pour l'adapter aux défis d'aujourd'hui et de demain, tant pour les entreprises que pour les salariés. Nous étions également tous conscients, lors de nos débats, de l'urgence d'agir,

la vivre. Aussi, l'accord obtenu en commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation, qui consacre des orientations pragmatiques, est le fruit d'un dialogue, à la fois au Parlement, mais aussi avec les partenaires sociaux, dans le cadre des concertations.

repose sur la confiance dans la capacité des partenaires sociaux, des employeurs, des salariés et de leurs représentants à trouver, par le dialogue, comment répondre aux besoins de liberté et de protection à la fois des entreprises et des salariés. Cela suppose un dialogue social renforcé, avec des acteurs responsabilisés et mieux formés, dans un cadre structuré, lisible et décentralisé. C'est ce qui permettra de trouver au plus près du terrain des solutions conciliant l'impératif de compétitivité et l'exigence de justice sociale, c'est-à-dire de faire converger l'économique et le social.

Je pense en particulier à la meilleure prise en compte de l'égalité femme-homme, mais aussi des personnes en situation de handicap. Je souhaite à ce propos remercier Mme la sénatrice Dominique Gillot d'avoir porté ces dispositions, qui ont ensuite été adoptées à l'unanimité. À ce stade, nous pouvons être collectivement satisfaits du résultat de cet alliage entre démocratie sociale et démocratie politique, sans préjuger les étapes ultérieures. Cet alliage a permis d'affiner utilement les orientations envisagées initialement par le Gouvernement. Je retiendrai plusieurs exemples où les débats ont fait évoluer notre conception du projet. Sur le premier volet, dédié à la nouvelle articulation de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche, ainsi qu'à l'élargissement sécurisé du champ de la négociation collective,

Elle transparaîtra dans la rédaction des ordonnances afin de garantir l'effectivité des droits pour tous les salariés et les employeurs, sans alourdir la charge administrative des entreprises. C'est tout l'esprit de la réforme du compte professionnel de prévention, qui allie justice sociale et simplicité pour les petites entreprises. Sur le deuxième volet, relatif à la clarification Sur le deuxième volet, relatif à la clarification des instances de représentation du personnel, vous avez été particulièrement sensibles à la nécessité de régénérer le dialogue social en introduisant une limitation du nombre de mandats syndicaux,

Aussi devons-nous renforcer davantage la formation mais aussi les parcours professionnels des représentants du personnel pour avoir un dialogue social de qualité et pour susciter des vocations afin de le faire perdurer. C'est l'objet de la mission que j'ai confiée à M. Simonpoli, président de l'association Dialogues, dont les recommandations auront vocation à trouver leur traduction dans les ordonnances. Vous avez également insisté sur la prise en compte de la spécificité de la taille ou du secteur d'activité des entreprises,

avec la même exigence qu'aujourd'hui. Enfin, sur le dernier volet, consacré à la sécurisation des relations de travail, outre l'accès simplifié au droit avec le code du travail digital, vous avez aussi approuvé les dispositions permettant de lever les incertitudes juridiques qui, de par leur caractère anxiogène, brident l'embauche. C'est l'enjeu de la sécurisation de la procédure de licenciement pour éviter le recours systématique au contentieux, néfaste tant pour l'employeur que pour le salarié, tous deux suspendus à des décisions de justice, parfois aléatoires, on l'a vu, ce qui les prive de se projeter dans l'avenir. C'est pourquoi nous souhaitons encourager la conciliation en amont, mais aussi augmenter les indemnités légales de licenciement, et clarifier le barème de dommages et intérêts.

sous l'oeil vigilant du législateur et des partenaires sociaux, mais aussi, à travers vous, mesdames, messieurs les sénateurs, de tous nos concitoyens. La mise en oeuvre de cette réforme et l'appropriation dont elle fera l'objet par les acteurs de terrain se fera en parallèle avec les prochains chantiers que le Gouvernement engagera ces dix-huit prochains mois pour rénover durablement notre modèle social. Je les ai déjà annoncés. Il s'agit de la réforme de l'assurance chômage, de la réforme la formation professionnelle, de la réforme de l'apprentissage que je défendrai avec le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il s'agit également de la réforme des retraites, que portera la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn. Cet ensemble de réformes, allié à l'action du Gouvernement en faveur de la compétitivité des entreprises et du pouvoir d'achat, doit permettre à la croissance, de retour dans l'Hexagone, d'être pleinement porteuse d'emplois,

Ces réformes interdépendantes constitueront le terreau sur lequel nos entrepreneurs pourront pleinement exprimer leur potentiel d'innovation, de création d'emplois et de promotion de l'excellence du savoir-faire et de la créativité de la France partout dans le monde. Plus de liberté et plus de protections grâce à un dialogue social renforcé au plus près du terrain, tel est le sens de la loi que j'ai l'honneur de soumettre à votre vote aujourd'hui. C'est l'esprit dans lequel nous engagerons les réformes à venir. Au terme de cette première phase du long chantier de rénovation que nous venons d'entreprendre, je souhaite remercier celles et ceux qui ont participé au débat. Je tiens tout particulièrement à saluer la rapidité et l'efficacité

Je tiens aussi à remercier, au nom de mon collègue Gérald Darmanin, le rapporteur pour avis sur l'article 9, Albéric de Montgolfier. Je souhaite par ailleurs saluer les présidentes et présidents de séance, qui ont permis que la discussion de ce texte se déroule dans de bonnes conditions et dans un très bon climat.

Je tiens enfin à saluer le travail remarquable et la disponibilité des administrateurs des commissions concernées, sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui. Enfin, je sais que le mandat de certains d'entre vous, touche à sa fin, ce qui vous privera de poursuivre nos échanges, en ce haut lieu de la République, sur la rénovation de notre maison commune que constitue le modèle social français. Pour autant, si vous n'avez pas la possibilité de revenir sur ces travées, je sais que votre engagement politique se poursuivra sous d'autres formes. Car nous sommes convaincus, même si nos points de vue diffèrent parfois, ce qui est le signe d'une démocratie vivante, que le modèle social français doit enfin être une réalité au quotidien pour l'ensemble des entreprises et de nos concitoyens. Car nous devons faire vivre la promesse républicaine de l'émancipation individuelle et collective, afin que chacun puisse se réaliser. C'est pourquoi nous rénoverons notre modèle social afin que la liberté d'entreprendre aille de pair avec le renforcement de l'égalité des chances, toutes deux fondements de la fraternité. Notre ambition commune, et je sais que vous la portez pleinement, c'est de faire en sorte que la France, forte de son héritage et de ses valeurs, puisse trouver et inventer en permanence sa propre voie vers un modèle social ambitieux et rénové, en phase avec les enjeux de notre temps, aujourd'hui comme demain. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, de moins en moins chers, d'ailleurs, la commission mixte paritaire a supprimé quelques amendements de la droite du Sénat, mais la mouture finale n'en reste pas moins marquée par des orientations très libérales simplification pour le chef d'entreprise afin de licencier plus facilement et moins cher, modifier les contrats de travail, exiger des sacrifices supplémentaires. C'est une grande régression sociale, car le salarié n'est pas seulement un producteur de richesse : c'est avant tout un citoyen qui a droit au respect de sa dignité, à la juste rémunération de sa contribution à la prospérité nationale et qui doit être un acteur du devenir de l'entreprise.

des latitudes nouvelles sont octroyées aux entreprises en détricotant les dispositifs qui protégeaient les salariés des abus, de l'arbitraire et de la précarité.

La dilution des CHSCT est un danger pour les salariés et, partant, pour l'entreprise. Vous dites offrir les mêmes compétences aux commissions. Comment y croire ? Il suffisait alors de conserver les CHSCT. limiter le nombre de mandats, alors que négocier face à un professionnel exige non seulement de maîtriser la matière juridique, les évolutions de carrière, le droit du travail, mais aussi d'apprendre sur le tas les stratégies, les écueils à éviter. La vertu n'inspire pas toujours chacun de nos citoyens. Vous dites « confiance ». C'est votre slogan maintes fois répété. Mais la confiance, ça se mérite. Croyez-vous que votre texte soit de nature à l'instaurer ? Les négociations collectives sans représentants syndicaux ni mandatement est la porte ouverte à tous les abus, toutes les pressions. C'est parce que, dites-vous, 96 % des PME-TPE n'ont pas de délégué syndical. Osons dire que, parfois, elles ne le souhaitent d'ailleurs pas. N'oublions pas qu'en cette période de chômage élevé une grande inquiétude étreint les salariés : 83 % d'entre eux craignent de perdre leur emploi, ce qui n'est pas sans conséquence sur les votes extrêmes. C'est dire si chacun d'eux se sent vulnérable et plutôt contraint à une certaine complaisance. Quelle valeur aura alors un accord d'entreprise accepté dans l'angoisse ? Il aurait eu une autre grandeur, madame la ministre, Il aurait eu une autre grandeur, madame la ministre, le défi que vous auriez pu vous lancer de favoriser le développement de la représentation syndicale. Mais vous faites l'inverse en lui déniant, dans les faits, toute utilité.

vous voulez la lui accorder pour des licenciements sans souci, l'élargissement du travail de nuit, des contrats de travail modifiés, des conditions dégradées. Le projet de loi va fabriquer de la précarité et de la régression sociale. La présomption de légalité de l'accord d'entreprise conduira le juge à restreindre son contrôle sur les accords collectifs. La réduction des délais de recours manifeste une volonté de limiter le nombre des victimes demandant réparation. Enfin, le plafonnement de l'indemnisation

Or les jugements étant individualisés, aucune situation ne ressemble à une autre. L'analogie avec la justice pénale est totalement injustifiée. Celle-ci prononce des sanctions contre les auteurs de délits.

la pénibilité. Vous introduisez une dichotomie regrettable entre les professionnels exposés, alors qu'il s'agit de la santé, de l'intégrité physique et mentale, de la durée de vie des ouvriers concernés. Vous abandonnez le choix de la prévention quand il s'agit de s'attaquer à la plus grande injustice qui soit. Les difficultés d'appréciation sont bien réelles, mais votre attitude est constante : la cause est juste, reconnaissez-vous, mais elle est difficile à satisfaire, alors abandonnons la cause.

l'idée que la généralisation des contrats de chantier invite les entreprises à l'utiliser en lieu et place du CDI : des millions de travailleurs précaires en France seraient alors privés d'accès au logement, aux banques, bref, de la sécurité du lendemain. A-t-on vraiment mesuré les effets toxiques de cette généralisation ? Pour justifier tous ces changements, vous chargez la France de tous les maux : ses charges sociales, ses rigidités, son incapacité à innover, à réagir.

Alors que les indicateurs économiques sont au vert, que la croissance repart, vous pensez que l'économie gagnera en vitalité par la dérégulation du marché du travail. Mais il ne peut y avoir de véritable croissance sans confiance en l'avenir, de la part des citoyens, des salariés, des entreprises, tous ensemble. Et la confiance dont vous avez bénéficié, j'ai peur que vous ne soyez en train de l'éroder au travers de ces mesures par trop déséquilibrées ! Vous voulez gagner la croissance en fragilisant les salariés. Vous récolterez la révolte des salariés et une économie, de nouveau, à la peine.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'encre de la loi El Khomri à peine sèche, le premier gouvernement Macron s'en inspire, s'engouffre dans la brèche et continue le démantèlement du code du travail, bousculant les « formidables garde-fous » dont l'ancienne ministre du travail nous avait tant vanté la solidité. La CMP a abouti. Quoi de plus naturel, en somme, qu'un accord entre une droite sénatoriale toujours aux avant-postes pour « libéraliser, toujours plus et une ministre du travail dont la conception de la « flexisécurité » se traduit par une corvéabilité accrue des salariés et une sécurité accrue pour les bénéfices, les stock-options des dirigeants et actionnaires Du dialogue social, notre ministre ne retient qu'une discussion au niveau de l'entreprise, là où le salarié est le plus faible face à l'employeur tout-puissant. En matière de cogestion, elle refuse que les salariés soient plus nombreux dans les conseils d'administration. Craignez-vous, madame la ministre, que si les travailleurs font la preuve de leurs capacités de décision au plus haut niveau, il ne soit plus possible de justifier les salaires de dirigeants cent fois plus élevés que le salaire moyen ? Vous l'aurez compris, mes chers collègues, les écologistes ne voteront pas ce projet de loi, cher au MEDEF, pris par le Gouvernement par ordonnances, au mépris de toute véritable négociation. Madame Bricq, remarquable idéologue du parti « en marche », ... Merci ! ... vous parliez, jeudi dernier, de l'importance de la formation professionnelle. Mais qu'a-t-on fait sous le gouvernement précédent, dont vous étiez déjà une émérite défenseure ? Pas assez ! J'ai proposé au Sénat, qui l'a votée à la quasi-unanimité en avril 2015, une résolution sur la mise en place d'un GPS pour l'emploi recensant les offres d'emploi non pourvues, analysant les causes pour proposer des solutions, en particulier en matière de formation. Qu'a fait ce gouvernement de cette proposition, madame Bricq ? Rien, rien de rien ! Quel gâchis ! collègues, c'est ma dernière intervention dans cet hémicycle où, je le reconnais, j'ai tant aimé débattre pendant les deux mandats que j'ai exercés. Je ne puis toutefois m'empêcher de ressentir un grand dépit quant à l'efficacité parlementaire. Le cadre de travail de notre institution est de haute qualité, à tous les niveaux, dans tous les services, de l'agent à l'administrateur principal. J'ai pu l'apprécier.

chers collègues, je vous souhaite, je nous souhaite une réforme en profondeur du fonctionnement de nos institutions. Sans cela, le discrédit du politique s'amplifiera, la déqualification du parlementaire perdurera.

monsieur le président-rapporteur, quand elle est conclusive. En effet, on dispose, pour une fois, d'une entière liberté, on est mis en face de sa responsabilité. Nous savons qu'il n'y a pas de mandat impératif pour un parlementaire. Il faut choisir la voie la meilleure pour arriver à un compromis positif. Quand on veut, on peut, et nous l'avons montré

Le quatrième point fort, qui est à mes yeux le plus important, c'est le renforcement du dialogue dans l'entreprise par la mise à niveau de la connaissance et de l'appréciation pour les salariés de la stratégie économique et sociale

réaffirmation de deux principes, celui des accords majoritaires, dont le calendrier de la généralisation est accéléré, et celui, ô combien important, de la présence syndicale.

était important. Pour le groupe La République en marche, notre objectif est atteint. L'exécutif, que nous soutenons fermement, garde sa latitude de réactivité aux propositions des partenaires sociaux

pour autant qu'ils retrouvent confiance en leur pays et en eux, car ils ont toute capacité pour être au premier rang.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'accord trouvé en commission mixte paritaire ne nous a pas surpris. La convergence d'idées sur ce texte entre la majorité sénatoriale et la République en marche avait été annoncée par le président Milon, dès l'examen en commission. Il avait déclaré ne pouvoir « qu'approuver la philosophie de ce texte » et « soutenir résolument la volonté du Gouvernement de libérer les entreprises des contraintes juridiques qui entravent leur développement Eh bien, c'est de cela qu'il faut continuer à débattre ! Car nous sommes ici au coeur de ce qui oppose la droite et la gauche, même si nous regrettons qu'une partie de cette dernière l'ait oublié en légitimant la loi El Khomri. Celle-ci posait pourtant les bases de la destruction du code du travail à laquelle on assiste aujourd'hui. Nous sommes fiers, au groupe CRC, de n'avoir pas faibli. Et nous serons toujours là, comme nous l'avons encore fait la semaine passée par la voix de notre présidente, pour rappeler les vérités qui fâchent ! Mes chers collègues, vous qui vous apprêtez à voter les conclusions de la CMP, pouvez-vous au moins nous expliquer en quoi les mesures annoncées dans ce projet de loi d'habilitation seront facteurs d'embauches et « de compétitivité de notre économie », comme l'affirmait aussi Alain Milon ?

c'est que si les Français s'opposent majoritairement à la philosophie de ce texte, ce n'est pas sans raison ! Ils ont en tête quelques épisodes peu flatteurs pour les partisans du libéralisme économique à tous crins. Qui ne se souvient pas, en particulier, de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui annonçait la création de 1 million d'emplois en contrepartie d'exonérations massives de cotisations sociales ? Les exonérations, elles ont été obtenues avec le CICE, mais où sont les emplois créés ? Croyez-vous vraiment que les mesures actées par la CMP iront dans le sens d'une modernisation de la démocratie sociale ? comparez-les aux conquêtes du Front populaire, à celles arrachées par nos prédécesseurs qui ont libéré la France et inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 que « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu'à la gestion des entreprises.

En réalité, vous inscrivez vos pas dans une offensive libérale, dont le seul but est de sacrifier les droits sociaux et démocratiques des travailleurs et d'empêcher toute action protectrice de l'emploi et des rémunérations, des conditions de travail et de santé dans chaque entreprise. Un progrès économique, la nouvelle formulation issue de la commission mixte paritaire, qui va permettre à des entreprises- cela a été rappelé -, alors qu'elles sont dans une situation économique florissante au niveau du groupe, de s'appuyer sur le périmètre national pour licencier massivement au seul profit des actionnaires ? Un progrès social, la réduction du délai de recours devant les prud'hommes en cas de rupture du contrat de travail ? Un progrès, la définition de plafonds obligatoires d'indemnisation des salariés victimes d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aujourd'hui une réparation intégrale du préjudice subi peut être obtenue Un progrès social et économique, la généralisation potentielle du CDI de chantier à de nouveaux secteurs d'activité, qui conduira à précariser ceux-là mêmes qui auront un CDI Un progrès, la nouvelle articulation des normes du droit du travail, qui aboutira à confier aux branches ce qui relevait jusqu'à présent de la loi- les contrats courts, par exemple -et affirmera la primauté de l'accord d'entreprise sur les normes conventionnelles et sur le contrat de travail On en connaît à l'avance les conséquences : le licenciement non économique pour un salarié qui refuserait une dégradation de ses droits, et un risque non négligeable de social orchestré par les grands groupes Rappelons-le, mes chers collègues, le code du travail est un outil de protection du salarié face à son employeur, pas un instrument d'amplification du chômage ou d'accélération de la rentabilité financière des entreprises. Et ce n'est certainement pas en retirant des droits aux salariés que vous résoudrez les difficultés, quant à elles très réelles, vécues par les entreprises, en particulier, les plus petites : l'incertitude économique, les délais de paiement, l'accès au crédit bancaire ou les difficultés à recruter du personnel qualifié et compétent. Oui, je le redis, il y a indigence à penser qu'une amélioration de la productivité pourrait résulter de la réduction des droits des salariés ! Quelle vision à courte vue ! Nous proposons exactement l'inverse, car l'entreprise est aussi un bien commun dont le développement durable nécessite l'adhésion et l'engagement de tous et, en premier lieu, de ceux qui produisent les richesses. Nous avons, au contraire, que votre projet s'adresse bien davantage aux patrons du CAC 40, qui réalisent des milliards d'euros de profit, qu'aux salariés dont le Smic ne sera pas revalorisé cette année. Le journal 'de ce jour explique comment les rémunérations complémentaires des dirigeants des grands groupes sont fondées sur le strict intérêt des actionnaires. C'est ainsi que huit des dix membres du comité de direction de Danone ont pu bénéficier de 4,8 millions d'euros de plus-values. indécent pour les salariés et leurs familles auxquels vous demandez en permanence des sacrifices ! Pour eux, pas de stock-options mais une force et une intelligence au travail qui doit au contraire être respectée et valorisée ! C'est ainsi que l'on améliorera l'efficacité économique et non en Notre combat n'est donc pas terminé. Il se poursuivra ici, dans l'hémicycle, lors de l'examen du projet de loi de ratification des ordonnances. Nous serons aussi présents le 12 septembre dans la rue, au côté des salariés et des syndicats qui s'opposent à ce projet de casse du code du travail, que nous rejetterons dans quelques instants par un vote unanimement contre du groupe communiste républicain et citoyen. Bravo ! La parole est à Mme Françoise Laborde. Madame la Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président-rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour entériner les conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue lundi après-midi. Si nous pouvons nous féliciter des débats constructifs et de l'adoption d'un texte commun, nous sommes plus circonspects quant à la méthode employée. Mon collègue Guillaume Arnell l'avait déjà souligné en première lecture, « les ordonnances constituent une forme de législation déléguée qui affaiblit le rôle du Parlement, au même titre qu'une interprétation trop restrictive du droit d'amendement ou le recours systématique à la procédure accélérée D'autant qu'il s'agissait, à l'origine, d'une procédure exceptionnelle, destinée à faire face à une situation urgente et pour un délai limité seulement. C'est la raison pour laquelle les sénateurs du groupe du RDSE sont réticents, je le répète, au fait de donner un blanc-seing au pouvoir exécutif, quel qu'il soit, surtout lorsqu'il s'agit d'une réforme d'une telle ampleur et que la concertation avec les partenaires sociaux se poursuit. Sur le fond, la majorité des membres du RDSE partagent les grandes orientations de votre réforme, qui vise à offrir plus de souplesse aux entreprises tout en protégeant les salariés. Nous devons en effet faire preuve de pragmatisme et adapter notre droit du travail à la réalité économique actuelle si nous voulons nous attaquer au chômage de masse que la France connaît depuis plus de trois décennies. pour nos concitoyens qui y sont confrontés, le chômage est une véritable souffrance : au-delà de la perte d'un salaire, le chômage constitue aussi la perte d'un lien social et une atteinte à l'estime de soi.

Alors, oui, inverser durablement la courbe du chômage est une impérieuse nécessité ! Lors de sa réunion, la commission mixte paritaire a confirmé plusieurs avancées proposées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je pense notamment au télétravail, à la suppression de la condition d'ancienneté minimale d'un an nécessaire à l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement, à la formation des représentants du personnel, à la prise en compte de la situation des personnes handicapées et de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore à l'exclusion de la barémisation des indemnités prud'homales pour les licenciements entachés par une faute de l'employeur d'une exceptionnelle gravité. S'agissant des points de divergence entre nos deux assemblées, les débats en commission mixte paritaire ont permis à nos collègues de dégager un consensus ; je m'en félicite. C'est le cas notamment de l'aménagement du calendrier de mise en place des accords majoritaires de la loi du 8 août 2016 auxquels nous sommes particulièrement attachés. C'est en effet la garantie de la légitimité des accords d'entreprise et des organisations syndicales. C'est le cas également de la réintroduction de la référence aux accords de maintien de l'emploi dans la liste des accords dont il est envisagé d'harmoniser le régime. Comme l'a rappelé le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, non seulement la suppression de la référence à ces accords ne suffisait pas à supprimer leur existence juridique, mais elle était, en plus, contre-productive puisqu'elle conduit à renoncer à l'harmonisation du régime juridique applicable aux accords de maintien de l'emploi avec les autres accords spécifiques mentionnés à cet alinéa. Je pense aussi à la mise en place obligatoire d'une commission exclusivement consacrée aux questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de la future instance unique de représentation du personnel. Si la CMP a conservé le caractère spécifique du motif de licenciement d'un salarié qui refuse l'application d'un accord collectif- tel que l'avait proposé notre commission des affaires sociales nous nous réjouissons qu'elle ait trouvé un compromis en proposant aux salariés un accompagnement spécifique sous la forme de droits complémentaires à la formation. S'agissant, en revanche, de l'encadrement des indemnités prud'homales, le groupe du RDSE est assez partagé, certains d'entre nous estimant que le barème indicatif mis en place par la loi El Khomri était suffisant. En revanche, nous nous félicitons de votre promesse de revaloriser le montant des indemnités de licenciement, qui, rappelons-le, sont parmi les plus faibles d'Europe. Madame la ministre, vous l'aurez compris, la majorité des sénateurs du RDSE soutiendra ce projet de loi d'habilitation, qui constitue la première étape de votre réforme. Pour autant, nous serons particulièrement attentifs aux mesures qui seront soumises à ratification dans quelques mois. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président-rapporteur de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, ce projet de loi d'habilitation permettant au Gouvernement de prendre par ordonnances des mesures pour le renforcement du dialogue social s'inscrit dans un objectif plus large de rénovation de notre modèle social. La modification du code du travail, l'allégement des contraintes supportées par les entreprises, la réorganisation des outils du dialogue social ne certes pas directement d'emplois- pas plus, d'ailleurs, que le CICE -, mais ils ont pour vocation de stimuler le désir d'entreprendre, d'investir et, au final, de favoriser le développement des entreprises et de l'activité économique dans notre pays. La création d'emplois est la conséquence de ce processus, qui s'inscrit dans un temps long, contrairement aux temps politique et médiatique qui ne sont souvent appréhendés que dans le court terme. La rapidité des évolutions technologiques, la révolution numérique, la multiplication des échanges financiers, économiques et humains représentent des bases factuelles d'un monde qui change et auquel nous devons permettre à notre économie et à nos entreprises de s'adapter. Tourner le dos à cette réalité et à ces évolutions dans un réflexe protecteur et protectionniste nous conduirait inévitablement sur la voie du déclin, avec toutes les conséquences néfastes que cela suppose sur le plan économique et social. Ce projet d'ordonnances est le prolongement de la loi du 8 août 2016, dite loi El Khomri, avec un champ d'intervention toutefois plus restreint. D'autres textes viendront compléter cette évolution, notamment en termes d'apprentissage, de formation professionnelle, d'assurance chômage et de retraite. à défaut d'une réécriture complète du code du travail, telle qu'elle avait été envisagée dans la loi El Khomri, il me paraîtrait indispensable de procéder à un toilettage simplificateur de ce code en supprimant nombre de dispositions inopérantes, complexes, qui ne relèvent pas toujours de la loi des précisions excessives qui pourraient venir limiter de manière trop contraignante le champ des négociations de branche ou d'entreprise. En ce qui concerne les domaines qui doivent être traités dans ces ordonnances, nous nous félicitons de la volonté du Gouvernement de prévoir des mécanismes opérationnels, c'est-à-dire qui pourront facilement trouver une traduction concrète dans la négociation sociale et le fonctionnement des entreprises. Il faut en effet éviter des dispositifs parfois fondés sur des intentions louables mais difficilement applicables, donc, peu utilisés. Je pense, en particulier, aux accords de maintien de l'emploi, les AME, que le Sénat souhaitait supprimer

Même si nous maintenons quelques réserves ponctuelles sur ce projet de loi, la version aujourd'hui soumise à notre approbation nous paraît satisfaisante dans les principales orientations qu'elle préconise. Nous sommes, en premier lieu, favorables aux modes de conclusions des accords d'entreprise, qui permettront d'en augmenter sensiblement le nombre, en particulier dans les PME et TPE, grâce à l'ouverture de ces accords, en l'absence de délégués syndicaux, aux délégués du personnel et en autorisant, en dernier ressort, une consultation directe des salariés. le périmètre à prendre en considération pour évaluer les difficultés d'une entreprise, même si ce dispositif mérite quelques

la fixation d'un barème obligatoire pour les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion d'un certain nombre de situations en raison de la responsabilité et du comportement de l'employeur. Nous approuvons, en le traitement différencié de certaines mesures pour les PME et TPE. Dans cette loi d'habilitation, le Gouvernement et vous-même, madame la ministre, avez fait preuve à la fois de pédagogie et de compréhension. L'Assemblée nationale et le Sénat, dans le respect du travail respectif de nos deux assemblées, ont su faire des concessions mutuelles et trouver un compromis équilibré pour présenter aujourd'hui un texte commun validé par la commission mixte paritaire. Nous nous félicitons du fait que de nombreuses propositions émanant du Sénat, de la commission des affaires sociales, en particulier, aient été retenues ou prises en compte dans la version finale. Nous le devons aussi à l'esprit très constructif dans lequel ont travaillé nos rapporteurs, que je tiens à féliciter. Le groupe Union Centriste et, j'en suis persuadé, une majorité de nos collègues se réjouissent de cette conclusion. Elle témoigne en effet d'une démarche positive du Parlement à l'égard de la procédure des ordonnances, qui aurait pu donner le sentiment de nous mettre quelque peu à l'écart. Nous souhaitons, bien entendu, que, conformément à l'article 8 de ce projet de loi d'habilitation, un débat puisse de nouveau s'engager avant la fin de l'année, le plus tôt possible après la promulgation des ordonnances, dans le cadre des lois de ratification. Madame la ministre, vous considérez ce texte comme « un pari sur la confiance dans le dialogue social ». Pour notre part, nous faisons aujourd'hui un pari sur la volonté du Gouvernement de simplifier et de rationaliser notre droit social. En votant le texte de la commission mixte paritaire, nous vous accordons notre confiance et nous formons le voeu, dans l'intérêt même de notre pays, qu'il s'agisse là de deux paris gagnants.

qu'il me soit permis de remercier le docteur Milon, président-rapporteur, pour ses commentaires toujours très pédagogiques. C'est l'homme de l'art au chevet d'un malade en crise, le chômage ! Je vous remercie également, madame la ministre, pour vos commentaires toujours très détaillés et courtois. Néanmoins, les ordonnances restent toujours une interrogation pour les parlementaires puisque les champs de propositions leur sont limités. Ils peuvent certes réduire le champ des ordonnances, mais pas l'élargir. Cette frustration a cependant été atténuée par les débats très ouverts que nous avons pu lancer sur nombre de sujets. Il faut dire que le groupe communiste républicain et citoyen nous a bien aidés Madame la ministre, c'est à l'efficacité de cette loi que l'on jugera de sa pertinence. Le débat sur la ratification des ordonnances et sur l'évaluation de ce processus législatif sera déterminant. Car la question est bien là : cette loi sera-t-elle efficace sur le plan de la compétitivité de nos entreprises, et surtout sur celui de la relance, tant attendue, En tout état de cause, on ne peut pas rester les bras croisés, compte tenu du taux de chômage qui caractérise notre pays par rapport aux autres États européens. Cette loi a au moins le mérite d'essayer de faire bouger les lignes ! Je voudrais rappeler trois faits essentiels

sociaux ni une atteinte à l'action des délégués du personnel ou des délégués syndicaux. C'est tout simplement une simplification pleine de bon sens, d'autant plus que la commission mixte paritaire a ouvert la possibilité à ces instances de créer des commissions spécifiques. Ce sera l'occasion de travailler au sein des entreprises sur les sujets essentiels, tels que les conditions de travail. C'est parce qu'elle prend en compte les préoccupations de ses collaborateurs qu'une entreprise peut être performante. C'est un facteur de gain de compétitivité essentiel et il n'y en a pas beaucoup pour nos entreprises, dont les charges sociales sont trop élevées dans ce pays. Le deuxième point important est le recours à la consultation. Cette possibilité offerte pour valider un accord, c'est le référendum d'entreprise, sur l'initiative des salariés, d'un syndicat représentatif ou de l'employeur. C'est une véritable avancée

-doivent permettre aux chefs de petites entreprises de ne plus refuser ces marchés ou de ne plus refuser d'embaucher. La balle sera dans leur camp.

Tous les territoires ne disposent pas du même débit nécessaire à la bonne marche de nos entreprises. Les propositions gouvernementales d'« un bon débit pour tous

Il est indispensable de poursuivre ce combat pour l'investissement dans le très haut débit fixe pour tous et pour toutes les entreprises de France. Votre loi pourra ainsi réussir encore mieux. L'égalité des chances pour chaque entreprise est aussi déterminante que l'égalité de nos concitoyens pour trouver du travail Madame la ministre, même si vous n'avez pas retenu toutes les propositions adoptées par la commission des affaires sociales du Sénat, sur l'initiative de son rapporteur- propositions toutes aussi pertinentes les unes que les autres -, je voterai ce texte avec le sentiment d'avoir essayé d'apporter une petite pierre à ce grand édifice qu'est la politique de l'emploi, laquelle, soit dit en passant, pourrait être décentralisée sur le plan régional. Bravo

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en cohérence avec l'appui apporté à la ministre Myriam El Khomri lors de l'élaboration de la loi Travail en 2016, j'exprime à nouveau, au nom de collègues du groupe socialiste et de moi-même, une approche favorable à la philosophie de ce projet de loi d'habilitation. Nous avons la conviction que, dans le monde mouvant d'une économie ouverte, de puissances financières insatiables, il existe pour la France une voie de progrès apportant aux salariés des protections nouvelles pour mieux construire leur vie professionnelle et armant nos entreprises pour affronter la concurrence mondiale. Madame la ministre, nous vous accompagnons quand vous affirmez que l'objectif est de renforcer le dialogue social. Nous avons néanmoins la conviction que cet objectif ne peut être atteint qu'en le liant étroitement au développement de la présence syndicale dans l'entreprise, des moyens donnés pour faire des syndicats les partenaires forts, responsables et incontournables du dialogue social. Ce projet doit être examiné dans un triple contexte. Le premier élément de ce contexte est notre protection sociale, que vous aborderez successivement à travers l'assurance chômage au champ élargi, l'apprentissage, la formation, qui est la première protection des salariés et la première obligation des entreprises, les retraites et le pouvoir d'achat. Notre modèle social, bâti sur le principe de solidarité, possède des valeurs profondes qui ne peuvent être remises en cause. Toutefois, malgré un engagement financier global de 750 milliards d'euros, il n'efface pas le cancer du chômage et la précarité dont sont victimes plusieurs millions de nos concitoyens. L'évolution, amorcée avec la loi El Khomri, vers des droits attachés à la personne plus qu'au statut peut être une réponse à l'impératif de mobilité de l'économie aujourd'hui. Le deuxième élément de contexte est la réponse à cette interrogation : que veut dire travailler de nos jours ? Quand la perte d'un emploi est une tragique perte d'identité, la question du sens du travail demeure permanente. Celui-ci s'épuise souvent dans son organisation. L'emploi introduit une contradiction lorsque le salarié ne peut s'approprier son outil de travail. N'ignorons pas, par ailleurs, les souffrances qui s'y déploient : suicide sur le lieu de travail, mises au placard, arrêts maladie successifs, procès, burn-out, épuisements ... Évidemment ! Le troisième élément, c'est la confiance des salariés à rétablir dans l'entreprise. La capacité d'un employeur et de ses salariés à trouver le meilleur compromis à leur niveau, au bénéfice de leurs intérêts respectifs, est trop souvent négligée. Le dialogue social, s'il ne suffit pas, n'en demeure pas moins un élément qui donne du sens au travail. Sans nier le lien de subordination, écartons l'idée que l'entreprise ne serait qu'un lieu d'oppositions et d'affrontements. J'en viens au texte lui-même. Plusieurs propositions de rédaction de l'article 1 adoptées par la commission mixte paritaire recueillent un avis plutôt favorable de notre part. Il en est ainsi de la réintroduction de la référence aux accords de maintien dans l'emploi, de la précision des droits à la formation renforcés dont bénéficierait un salarié refusant de se voir appliquer les stipulations d'un accord spécifique, de la précision que le pouvoir de modulation du juge doit tenir compte aussi de l'intérêt des salariés, de la généralisation progressive des accords majoritaires, dont l'objectif est de renforcer la légitimité des accords d'entreprise. Nous marquons, en revanche, notre opposition au recours à la consultation des salariés pour valider un accord sur la seule initiative de l'employeur. Sur l'article 2, recueillent un avis plutôt favorable de notre part : la nouvelle rédaction de la fin de l'alinéa 2 définissant les conditions dans lesquelles une commission spécifique traitant des questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être créée au sein de l'instance unique le fait de ne pas déléguer systématiquement, sauf accord contraire, la compétence de négociation aux représentants des salariés en présence d'un délégué syndical ; le rétablissement d'une disposition relative à l'amélioration des conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d'administration et de surveillance des entreprises. Sur l'article 3, nous sommes plutôt favorables à la suppression, introduite au Sénat, de l'obligation de réduire d'au mois de moitié le délai de recours en cas de rupture du contrat de travail. Nous demeurons opposés à l'instauration d'un plafond et d'un barème aux dommages-intérêts accordés par les conseils de prud'hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Nous sommes sensibles, en revanche- et nous attendons la suite ! -, à l'introduction d'éventuels aménagements à la règle s'agissant de la prise en compte du périmètre national par le juge pour l'appréciation du motif économique, ce qui doit permettre de garder la prérogative d'appréciation du juge et d'éviter que des entreprises n'inventent des difficultés artificielles pour licencier. Madame la ministre, au regard de ces éléments, notre jugement définitif se forgera lorsque nous prendrons connaissance de la rédaction des ordonnances. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur et président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, notre groupe, bien que regrettant la procédure employée par le Gouvernement, approuve l'essentiel des principes exprimés dans le présent texte. Depuis plusieurs années, en effet, nous appelons à simplifier l'environnement juridique des entreprises, qui représente trop souvent un frein à leur développement, et donc à l'emploi. Le projet de loi présente un ensemble de dispositions allant dans ce sens. Nous en avons d'ailleurs déjà présenté certaines lors de l'examen des lois Macron, Rebsamen ou El Khomri. Il en est ainsi de la rationalisation des institutions représentatives du personnel, de la reconnaissance juridique des accords de flexisécurité, de la création d'un référentiel obligatoire pour fixer les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui va enfin permettre d'harmoniser celles-ci, ou encore de la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité, dénoncé pour sa lourdeur par l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. En outre, nous avons fait en sorte de préciser le texte, qui entretenait un certain flou sur des points importants. Ce flou, inhérent à la procédure d'habilitation, a permis au Gouvernement d'ajuster son texte en tenant compte des réactions que celui-ci a suscitées. Or, bien qu'il soit important de prendre en considération le résultat des concertations menées menées avec les partenaires sociaux, il nous semble que l'ambition initiale risque de sortir amoindrie des discussions menées avec eux. Je me réjouis donc que notre Haute Assemblée ait pu renforcer le texte sur plusieurs points essentiels et prendre ainsi quelques assurances quant à la future orientation des ordonnances. À la suite de notre rapporteur, je voudrais rappeler ces sujets qui nous semblent particulièrement importants. Tout d'abord, je me réjouis de la possibilité donnée à l'employeur de proposer un vote à ses employés sur des dispositions n'ayant pas obtenu l'aval des syndicats majoritaires. Certes, madame la ministre, vous n'étiez pas hostile à cette mesure, mais elle ne figurait pas clairement dans le projet de loi, qui prévoyait seulement de « faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord S'il s'agit de favoriser le dialogue social dans l'entreprise de manière concrète, par référendum, il faut l'écrire clairement, ce qu'a fait notre président-rapporteur. étant particulièrement à l'écoute des petites entreprises, je me réjouis par ailleurs qu'une solution ait été trouvée pour permettre des négociations, même en l'absence de représentation syndicale, avec les élus du personnel ou avec les salariés mandatés. Autre point introduit par le Sénat, qui me semble très important aux yeux des investisseurs : le choix du périmètre au niveau duquel le juge pourra apprécier les difficultés économiques d'une entreprise devant licencier. Un temps envisagée par le précédent gouvernement, la référence à un périmètre « national » a fait débat, avant d'être retirée du projet de loi de la ministre Myriam El Khomri, ce qui a contribué à l'insécurité juridique ressentie par les entrepreneurs sur notre territoire. Aussi avons-nous tenu à inscrire ce principe dans le présent texte, en laissant toutefois au Gouvernement la possibilité de déterminer d'éventuels aménagements à cette règle. J'évoquerai encore certains sujets importants. Nous avons encadré le fonctionnement de l'instance qui fusionnera les IRP, en fixant le nombre maximal des mandats qui y seront exercés, en renforçant la transparence de ses comptes ainsi que les règles de concurrence en cas de recours à l'expertise. Nous sommes parvenus à un accord en commission mixte paritaire pour maintenir la capacité de l'instance à participer aux négociations de l'entreprise. Nous regrettons cependant que celle-ci ne soit pas reconnue d'office et dépende d'un accord collectif. Notre satisfecit n'empêche d'ailleurs pas les mises en garde. Nous ne souhaitions pas, par exemple, revenir sur le sujet de la représentation des salariés au sein des conseils d'administration, déjà débattu lors de la loi Rebsamen. Les députés ont souhaité maintenir cette mesure dans l'habilitation, que nous avons pu, cependant, encadrer il ne sera pas question de revenir sur les seuils qui ont déjà été modifiés. Et nous avons précisé que les modifications apportées par le Gouvernement devront porter sur la formation des salariés. Autre point, nous n'avons pas pu maintenir un licenciement en cas de refus d'un accord collectif par un salarié, mais nous avons obtenu que ce licenciement ne soit pas non plus qualifié en licenciement économique, ce qui aurait créé de lourdes contraintes pour l'entreprise. Nous souhaitons le meilleur accompagnement possible pour les salariés, mais nous veillerons à ce que les règles fixées par ordonnance ne renforcent pas les contraintes pesant sur les entreprises. Je dirai ensuite un mot sur un débat que le Gouvernement a souhaité rouvrir, celui de la généralisation des accords majoritaires. Nous avons contesté cette règle créée par la loi Travail, car elle risque de bloquer le dialogue social dans les entreprises. Elle a d'ailleurs été fortement décriée par de nombreux intervenants entendus en audition. Nous manquons de recul sur l'application du dispositif, et il ne nous semble pas bien venu d'accélérer sa mise en place. La rédaction de compromis trouvée en a permis de supprimer le terme de « généralisation », mais a toutefois maintenu une habilitation du Gouvernement à « aménager le calendrier et les modalités de généralisation de ce caractère majoritaire ». Nous serons très vigilants sur la rédaction de l'ordonnance concernée. Nous parvenons, au terme de l'examen de ce projet de loi d'habilitation, à l'annonce de mesures que nous soutenons, mais, vous l'aurez compris, avec certaines réserves. Nous examinerons donc avec attention le projet de loi de ratification des ordonnances, qui, je l'espère, nous sera rapidement présenté, une fois les négociations sociales achevées. Enfin, ne nous leurrons pas, bien que globalement intéressantes, les mesures envisagées ne sont qu'un premier pas pour créer une véritable dynamique et relancer l'emploi. Des sujets essentiels que nous avons proposés en séance, comme la fixation par accord de la durée hebdomadaire du travail, le recours au temps partiel ou le relèvement des seuils sociaux, restent absents du projet de loi, dont le périmètre ne peut être élargi. J'ai également la conviction que seules des réformes structurelles et un allégement de la réglementation sociale relanceront la dynamique de l'emploi dans notre pays. En conséquence, le groupe Les Républicains votera le texte issu de l'accord intervenu en commission mixte

après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Personne ne demande la parole ?

Merci